Pourtant, depuis plusieurs années, on constate la disparition régulière des pharmacies dans les zones à faible densité géographique. La France est même passée sous le seuil des 20 000 pharmacies d’officine en 2023. Ce phénomène, qui touche essentiellement la profession de pharmacien titulaire, s’explique notamment par la restructuration du maillage officinal, marqué par le regroupement croissant d’officines. L’âge moyen du pharmacien d’officine est désormais de 46,7 ans, et il augmente petit à petit du fait de l’allongement des carrières.

Dans les grandes villes, dont beaucoup sont surdotées, la suppression de pharmacies par restructuration ne prête pas forcément à conséquence. En revanche, cette évolution est très préoccupante dans les petites communes, qui, bien souvent, ont déjà vu partir le médecin généraliste.

Les difficultés d’accès aux pharmacies sont d’autant plus problématiques que de nouvelles missions, destinées à améliorer l’accès aux soins des patients, ont été confiées aux pharmaciens d’officine au cours des dernières

plus de six ans après sa publication, le décret nécessaire à son application n’a toujours pas été pris. Pour nous, élus du groupe RDPI, la lutte contre l’apparition de déserts pharmaceutiques ne peut plus attendre. Néanmoins, nous ne sommes pas favorables à la modification des critères de droit commun d’ouverture des pharmacies d’officine choix qu’opérait le texte initial, au risque de déstabiliser inutilement le réseau existant. Nous saluons donc l’équilibre trouvé en commission des affaires sociales pour rendre les dispositions relatives aux territoires fragiles applicables, au plus tard, le 1 octobre 2024.

Chacun a pu le constater, si besoin était, au plus fort de la lutte contre la pandémie de covid 19 : les pharmaciens se sont alors mobilisés au service de la population. Dans notre pays, le nombre de pharmacies d’officine diminue de manière constante et préoccupante depuis maintenant dix ans. En résulte une baisse significative de la densité des officines.

Il nous faut donc agir. On peut déplorer que deux dispositifs législatifs destinés à préserver l’approvisionnement en médicaments des territoires les moins bien dotés demeurent à ce jour inappliqués. Pour maintenir l’accès aux médicaments dans les communes à très faible population, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique de décembre 2020 a autorisé, à titre expérimental, la création d’une antenne d’officine par un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’une commune limitrophe, lorsque la dernière officine de la commune d’accueil a cessé son activité et que l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population y est compromis.

fragiles, où l’accès aux médicaments n’est pas assuré de manière satisfaisante. Au sein de ces territoires, l’ouverture d’une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est possible lorsque celle ci est située dans un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine, sous deux conditions démographiques

et déjà prévus par la loi. L’ouverture de pharmacies d’officine dans les communes rurales sera ainsi facilitée et des aides pourront être octroyées pour favoriser leur maintien.

Je veux remercier

Depuis 2012, nous avons perdu 2 000 pharmacies, alors que notre population a augmenté de 4 % et que les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 20 % de nos concitoyens. En dix ans, nous avons perdu quatre officines pour 100 000 habitants, soit la plus forte baisse des pays de l’OCDE.

Monsieur le ministre, lorsque le Gouvernement agit de la sorte avec la santé des Français, on parle non plus seulement de dysfonctionnement, mais aussi de mépris. Il est plus que jamais nécessaire que le Gouvernement se ressaisisse et répare ces deux points majeurs.

depuis plusieurs années ou parfois plus récemment, ils dépistent, vaccinent et peuvent même traiter certaines pathologies bénignes. Dans tous les cas, ils entretiennent un lien humain avec leurs patients, pour lesquels ils sont de véritables interlocuteurs de confiance. est peut être encore plus vrai aujourd’hui dans certaines communes rurales, où il est parfois plus simple de s’adresser au pharmacien que de réussir à trouver un médecin.

À cela s’ajoute la question de l’attractivité des petites communes, sans oublier la place des pharmacies dans l’écosystème de la vie économique et leur importance dans le lien social. L’épidémie de covid 19 a d’ailleurs mis en évidence qu’il est important de disposer d’un maillage territorial d’officines suffisamment dense pour répondre aux situations de crise. Néanmoins, force est de constater que, chaque mois, vingt cinq pharmacies ferment en France. Entre 2007 et 2023, notre pays a perdu 4 000 officines. Cette situation reste préoccupante dans les petites communes, dont les habitants ont bien souvent déjà vu leur médecin généraliste

raisonnable pour l’ouverture d’une deuxième officine, car la tranche de 4 500 habitants reste trop contraignante. Par ailleurs, les conditions démographiques sont appréciées sur une durée au moins égale à deux ans. Là encore, ce critère est trop contraignant, notamment lorsque l’évolution démographique est avérée ou prévisible. J’avais aussi dénoncé certaines pratiques liées à l’acquisition d’officines. En effet, des pharmaciens profitent de la mise en vente d’une officine voisine concurrente pour l’acheter dans le seul but de faire cesser son activité. Face à de telles pratiques, les élus locaux, principaux acteurs de la dynamique territoriale, demeurent désemparés, même si la population de leur commune augmente. Il conviendrait de mieux encadrer ces procédés. En outre, il est essentiel de prendre en compte l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des besoins de santé de nos concitoyens, qui souffrent à la fois du manque de professionnels de santé et de la pénurie de certains médicaments.

Dans ce contexte, nous tenons à saluer cette proposition de loi visant à faciliter l’ouverture d’officines dans les territoires faiblement peuplés au moyen de transferts, de regroupements ou de créations.

L’idée est simple : recentrer le dispositif sur sa cible prioritaire. Cet amendement tend ainsi à contraindre le Gouvernement à publier, avant le 1 octobre 2024, le décret nécessaire à l’application du dispositif Territoires fragiles, qui prévoyait l’assouplissement des conditions d’ouverture des pharmacies d’officine dans les zones les moins bien

et des particularités géographiques de chaque zone. Dans ces territoires fragiles, l’ouverture d’une officine est facilitée dans une commune de moins de 2 500 habitants. Elle peut être autorisée si celle ci est située dans un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine, lorsque l’une d’elles recense au moins 2 000 habitants et lorsqu’elles totalisent ensemble au moins 2 500 habitants. Enfin, des aides spécifiques peuvent être accordées par l’ARS ou l’assurance maladie aux officines situées dans ces territoires pour favoriser leur ouverture et leur maintien. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte. La parole est à M.

tests médicaux, vaccinations, prescriptions médicales, télémédecine ou tout simplement conseils de santé délivrés à ceux qui ne peuvent aller chez un médecin. Avec la multiplication des déserts médicaux, les pharmaciens sont de plus en plus sollicités pour compléter l’offre de santé.

des problèmes de conflit d’intérêts et souvent de pérennité, auxquels il est utile de remédier. Ainsi, cette proposition de loi est positive pour nos concitoyens ruraux, qui ont droit à des services de santé de qualité et de proximité. Ce débat illustre la nécessité de réglementer l’installation des professionnels de santé sur les territoires. Si les critères d’installation doivent parfois évoluer, l’encadrement par la loi de la répartition territoriale des pharmaciens

que celles ci relocalisent leurs usines. Nous devons avoir des garanties concrètes d’emploi et de production. Dans cette optique, nous avions soutenu la création d’un pôle public du médicament et des produits de santé, sur l’initiative de nos collègues du groupe CRCE K. Nous soutenons cette proposition de loi et vous appelons, mes chers collègues, à adopter les amendements

Dans le contexte de la désertification médicale et du recul des services publics hospitaliers ou de maternité, la présence d’une pharmacie est devenue indispensable pour nos concitoyens, qui peinent à accéder aux soins.

les petites communes en modifiant le seuil à partir duquel il est possible d’ouvrir une officine. La réglementation actuelle pénalise les communes de moins de 2 500 habitants, qui ne peuvent ouvrir une officine de pharmacie sans se regrouper avec une autre commune comptant au moins 2 000 habitants. La commission des affaires sociales a préféré appliquer le dispositif

dépistages, vaccinations – et bientôt dans la prescription pour certaines maladies – je pense à l’angine et à la cystite. L’élargissement de ses missions est bien perçu par la profession, qui considère tout de même

de pharmacie. En effet, si l’on constate une baisse du nombre de primo inscrits au tableau de l’ordre des pharmaciens, on note aussi que 1 027 places ont été perdues en deuxième année de cursus en 2022 2023.

je suis persuadée que les défis de la formation et de l’attractivité demeurent essentiels.

cette proposition de loi, qui vise à maintenir l’accès à une pharmacie dans les communes les plus rurales, révèle parfaitement un grand mal français : les textes inappliqués. En effet, le dispositif Territoires fragiles, créé par l’ordonnance du 3 janvier 2018, prévoit déjà l’application de conditions d’ouverture assouplies dans les zones les moins bien dotées. Toutefois, il demeure inappliqué. Rendez vous compte : plus de six ans après la publication de l’ordonnance, le Gouvernement n’a toujours pas publié le décret nécessaire ! Ainsi, on peut toujours, autant qu’on le souhaite, se réjouir de l’adoption d’une nouvelle loi ou, en l’occurrence, de la publication d’une ordonnance, mais s’il manque le décret d’application, elle reste une coquille vide, un coup d’épée dans l’eau, un effet de manche, une vulgaire opération de communication. Nous sommes nombreux à parcourir nos départements ; or, mes chers collègues, du fait de ces textes inappliqués, vous percevez comme moi le découragement d’un grand nombre d’élus. De cette perte de confiance à l’égard de l’action publique découle une défiance à l’encontre du personnel politique. Nous devons en prendre toute la mesure, afin de lutter contre l’abstention, certes, mais aussi contre ceux qui souhaitent instrumentaliser cette colère légitime à des fins bassement électoralistes. Face à ce constat, le Parlement, je le conçois parfaitement, peut être tenté de se substituer au pouvoir exécutif. Ce faisant, il contribuerait à alourdir encore un peu plus notre droit, qui est, rappelons le, parfois bien difficile à rendre lisible. Pour lutter contre ces textes inappliqués, car inapplicables, nous devons plutôt choisir de nous investir pleinement dans notre rôle de contrôle de l’action du Gouvernement. En la matière, permettez moi de souligner ici l’important travail réalisé au sein de notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont j’ai le plaisir d’être membre. Ainsi, s’agissant de cette proposition de loi, en commission des affaires sociales, nous avons adopté le texte réécrit sur l’initiative de Mme la rapporteure, dont je salue le travail de synthèse et d’équilibre. Désormais, le texte contraint le Gouvernement à publier, avant le 1 octobre 2024, le décret nécessaire à l’application du dispositif déjà prévu. Dans le cas contraire, il appartiendra aux directeurs des ARS, à compter de cette date, d’identifier les territoires fragiles de leur ressort, sur la base des seuls critères légaux, et d’appliquer en leur sein les conditions d’ouverture assouplies devant favoriser, vous l’aurez compris, l’installation de pharmacies d’officine. Si la France a perdu plus de 1 800 pharmacies entre 2012 et 2022, alors que sa population augmentait de 3,7 %, il revient aujourd’hui au Gouvernement de prendre ses responsabilités afin de protéger ce maillage territorial. Dans un contexte accru de désertification médicale, il est primordial de veiller à assurer l’accès à une pharmacie dans les communes rurales. Je pense notamment, bien sûr, à mes Cévennes gardoises. Monsieur le ministre, soyez assuré que le Sénat y veillera

Elle a ainsi souhaité entendre les inquiétudes des pharmaciens, qui craignent qu’une révision des critères de droit commun d’ouverture des pharmacies d’officine applicables à l’ensemble du territoire national ne déstabilise profondément le réseau existant. Le dispositif Territoires fragiles apportera une première réponse dans les zones qui connaissent le plus de difficultés.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

De telles dérogations, lorsqu’elles étaient permises dans les années 1980 et 1990, ont donné lieu à l’ouverture d’officines aujourd’hui peu rentables et souvent amenées à fermer. Tous les représentants de la profession que j’ai rencontrés lors des auditions ont jugé une telle prérogative dangereuse pour le réseau. L’avis de

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aude, Cantal, Côte d’Or, Côtes d’Armor, Drôme, Eure et Loir, Finistère, Gard, Indre, Indre et Loire, Isère, Jura, Loir et Cher, Lot, Lozère, Marne, Haute Marne, Morbihan, Orne, Pas de Calais, Pyrénées Atlantiques, Sarthe, Haute Savoie, Var et Tarn

Les médecins propharmaciens ne sont pas une survivance du passé. Ils sont l’une des solutions dont nous disposons pour faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir un accès aux médicaments dans de bonnes conditions.

vocation est de traiter les patients dans leur environnement et non de délivrer des médicaments prescrits par d’autres professionnels de santé. Il n’est pas non plus souhaitable d’autoriser les infirmiers à délivrer des médicaments prescrits par les médecins